Je pense que nous ne sommes pas la voiture-balai du Parlement français. Dans ce cadre, l'absence de M. Véran, quasi permanente, y compris ce matin lors de la nouvelle lecture du PLFSS,

On vous aime bien, parce que vous êtes là, que vous prenez du temps pour travailler avec nous et que vous prenez le soin de respecter la représentation nationale. Vous agissez cependant dans une logique de solidarité gouvernementale

cette élasticité a des limites en pleine période budgétaire, surtout lorsque nous discutons de dépenses exceptionnelles, dans leur nature comme dans leur montant. Sans rien enlever à la compétence des représentants du Gouvernement présents depuis le début de l'examen de saluer le ministre Olivier Dussopt -ni au respect que nous avons pour eux, il ne nous semble pas acceptable de n'avoir que trop rarement l'honneur de la présence du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; relance dont nous allons précisément discuter dans quelques instants. Le Sénat est non pas une instance consultative, mais une assemblée parlementaire de plein exercice, chargée, entre autres, d'autoriser la perception des impôts et de voter la loi de finances. À ce titre, il nous paraît indispensable, durant cette période si particulière qui engage fortement nos finances publiques, que le ministre chargé des finances vienne expliquer les choix du Gouvernement et débattre avec la représentation nationale. Rendez-nous visite, monsieur le ministre de l'économie : cela nous ferait plaisir

en effet, de la considération pour vous : vous avez accepté d'intervenir devant mon groupe, nous discutons volontiers avec vous et vous discutez volontiers avec nous, vous répondez à toutes les questions et le faites avec courtoisie on vous aime bien ! Peut-être pourriez-vous devenir ministre de l'économie et des finances

Nous commençons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits des missions « Plan

et préserver, autant que faire se peut, le droit de chacun à présenter ses amendements. Enfin, je vous rappelle que nous devons achever l'examen de cette mission et de l'ensemble des articles rattachés, ce soir, à minuit et demi.

d'une demande d'examen séparé des amendements portant sur les crédits de la mission « Plan de relance », à l'exception des amendements portant sur un même sujet,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les missions « Plan de relance » et « Plan d'urgence face à la crise sanitaire ». Cette dernière mission ne comporte, toutefois, à l'heure qu'il est, aucun crédit pour 2021. Or cette mission, nous le savons d'ores et déjà, récupérera des crédits importants reportés de 2020 sur les différents dispositifs d'urgence. Le Gouvernement a même indiqué qu'il demanderait l'ouverture de crédits budgétaires supplémentaires. Je regrette que cela ne soit pas réalisé dès l'examen du PLF au Sénat, alors que le Président de la République s'est exprimé

Peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, nous donner des informations sur ce point. Je parlerai davantage, cet après-midi, de la mission « Plan de relance », qui déroge largement aux principes budgétaires, notamment à celui de la spécialité des crédits, puisqu'elle abonde des politiques publiques très variées. Elle comprend trois programmes tellement vastes que, par application du principe de fongibilité, l'autorisation parlementaire laissera une grande liberté d'action aux gestionnaires de programme. programme. Cette mission, avec 36 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et 22 milliards d'euros de crédits de paiement, ne représente qu'un peu plus du tiers des 100 milliards d'euros présentés par le Gouvernement comme périmètre du plan de relance.

Ce plan de relance constitue donc, avant tout, un plan de rattrapage pour des actions que les ministères auraient dû déjà conduire, et qui, dans la mission « Plan de relance », trouvent un véhicule budgétaire d'opportunité. Lorsque des dépenses portent sur le fonctionnement ou sur des achats courants, l'impact, en termes de relance de l'économie, est en effet pour le moins douteux. Nous aurons souvent le sentiment, aujourd'hui, de discuter un budget en réduction et d'anticiper sur les débats qui seront consacrés aux missions budgétaires dans les jours à venir. L'hétérogénéité de cette mission amène à s'interroger sur son objectif. Le dispositif traditionnel des objectifs de performance budgétaire est trop limité pour couvrir l'ensemble des politiques concernées. Le seul objectif clairement identifié et répété par le Gouvernement est la volonté de consommer les crédits rapidement : tel est, en effet, l'objectif fixé aux responsables de programmes, aux préfets et aux porteurs de projet. Or je crains que le Gouvernement ne confonde parfois la rapidité de consommation du budget, d'une part, et l'efficacité de mise en oeuvre concrète des projets, d'autre part. Pour que nous soyons vraiment dans les temps de la relance, il aurait fallu, comme le Sénat l'avait préconisé cet été, On risque aujourd'hui de favoriser des projets plutôt faciles à mettre en place, au détriment de projets plus structurants et plus durables, qui également, portent fortement l'empreinte de l'écoresponsabilité. C'est pourquoi, afin de rattraper le retard accumulé et de pouvoir afficher des résultats, le Gouvernement multiplie, en ce moment, les appels à projet et les appels à manifestation d'intérêt, alors que les entreprises sur le terrain témoignent du fait qu'elles ne sentent toujours pas les effets il y aura encore de nombreuses étapes d'ici à ce que la création d'activités se concrétise dans les territoires. Je ne pense pas que l'organisation que le Gouvernement est en train de mettre en place rapproche véritablement les sommes importantes, versées dans le plan de relance, des personnes, des entreprises et des acteurs qui devraient en bénéficier. Au lieu de véritablement travailler en partenariat avec les collectivités et leurs élus, qui connaissent bien leur territoire, en particulier avec les régions qui ont la compétence économique et conduisent une stratégie de développement, le Gouvernement met en place une organisation trop verticale. Les principaux dispositifs sont mis en oeuvre de manière uniforme au niveau national : je pense par exemple à la réforme des impôts de production, aux aides « de guichet » comme MaPrimeRénov'ou aux appels d'offres des grands opérateurs. Quant aux dispositifs qui peuvent être mis en oeuvre localement, ils sont très centrés autour des préfets, lesquels rendent compte au ministère de l'économie, attribuent les enveloppes en fonction des critères fixés à l'échelon national et font remonter l'information vers le ministère.

Malgré les insuffisances de ce plan de relance, il n'en reste pas moins que l'aide apportée dans les mois à venir sera décisive : alors que nous alternons entre des phases de confinement et de déconfinement partiel, il est indispensable, aujourd'hui encore plus qu'hier, de donner une visibilité, même imparfaite, sur l'action de l'État. Je présenterai au nom de la commission certains amendements tendant notamment à améliorer le ciblage du plan de relance sur les mesures qui me semblent les plus efficaces. Je soutiendrai également certaines des propositions faites par les membres de notre assemblée. Il faut en effet renforcer les politiques de l'emploi, en particulier pour les travailleurs jeunes ou peu qualifiés, qui sont les premiers à souffrir de la crise. Le fonds de solidarité devrait également évoluer. À cet égard, j'ai bien entendu les annonces du Président de la République, mais elles n'ont pas encore été traduites dans les textes et je reste persuadé qu'il faut travailler à une aide couvrant les charges fixes, y compris pour ceux qui ne subissent pas actuellement une fermeture administrative. Enfin, je vous proposerai d'augmenter le budget de la prime à la conversion et d'apporter des aménagements aux contreparties demandées aux entreprises bénéficiant des crédits de la mission.

Nous demandions au ministre de l'économie, des finances et de la relance un rapide effort de soutien et de relance économique et nous lui transmettions de nombreuses propositions en ce sens. Dès le mois de juin, la commission des affaires économiques du Sénat lui adressait son plan de relance. Cinq mois plus tard, le Sénat est appelé se prononcer sur la copie du ministre, traduction budgétaire du plan France Relance. Or la France n'est déjà plus la même. Alors que, en septembre, un fort rebond se dessinait, en novembre, l'économie est de nouveau figée par un second confinement, qui fait peser une menace existentielle sur notre petit commerce, frappe de nombreux secteurs et met à l'épreuve notre système social. Même les secteurs dont l'activité est relativement préservée craignent désormais un ralentissement durable. Face à l'incertitude, une crise de la demande vient remplacer la crise de l'offre.

la numérisation et la transition énergétique, le renforcement de notre souveraineté industrielle dans les secteurs stratégiques et l'enjeu d'innovation et de développement des compétences. L'effort budgétaire consenti est considérable. La commission des affaires économiques invite toutefois à rééquilibrer ce plan. À trop viser la France de 2030, on en oublierait la France de 2021 ; or le stimulus doit être au rendez-vous. La mission néglige d'importants leviers de relance et des angles morts

La mobilisation des crédits dès 2021 sera trop limitée, une partie importante d'entre eux allant vers des politiques de long terme, à l'effet d'entraînement incertain. À l'inverse, les chiffres annoncés pour la mission « Plan de relance » sont gonflés par le transfert purement cosmétique de crédits relevant du plan d'urgence ou de financements ordinaires.

ces carences impliquent que le Gouvernement fasse un effort particulier en termes de suivi et d'évaluation, sous le regard vigilant du Parlement. Sous ces réserves, que nous avons traduites en amendements, la commission des affaires économiques du Sénat-

Les premières ont d'ores et déjà été concrétisées en euros sonnants et trébuchants, les secondes manquent encore de matérialité. En fait, les mesures de sauvetage et les mesures de relance forment un continuum de l'action publique au service de notre économie et de son nécessaire redémarrage. Cette nouvelle mission constitue un outil comptable indispensable au travail du Parlement, qui pourra ainsi suivre l'affectation et la bonne utilisation des crédits votés, puis, le moment venu, évaluer leur performance.

Le second, c'est la fongibilité des crédits contenus dans les trois programmes de la mission. La combinaison de ces deux éléments doit garantir une exécution efficace des crédits de la mission dans un temps limité, sans doute trop limité. Le plan de relance est nécessaire ; surtout, il doit faire l'effet d'un électrochoc sur notre économie. Cette intensité d'exécution ne doit pas nous empêcher de préparer les fondements d'une croissance renouvelée-

Je tiens à cet égard à évoquer les deux leviers d'action qui me paraissent les plus efficaces. Le premier, c'est la rénovation énergétique de nos logements. Actionner ce levier nous permettra, d'une part, d'atteindre enfin les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour ce secteur qui demeure l'un des plus énergivores et des plus émetteurs de gaz à effet de serre,

Les collectivités territoriales doivent prendre toute leur part dans cette dynamique d'investissement. Les élus locaux sont sans doute les mieux placés pour organiser au plus près du terrain la mise en oeuvre de ce nécessaire élan national. C'est pourquoi je soutiens les amendements de Mme la rapporteure des affaires économiques qui cherche à provoquer un électrochoc à la fois sur l'offre et sur la demande. Je regrette que le Sénat n'ait pas pu, à ce stade, accepter le taux réduit de TVA sur les opérations de rénovation. J'espère que nous adopterons ce taux sur les capacités d'investissement des collectivités. Le second levier d'action, c'est le développement des énergies d'avenir, au premier rang desquelles figure l'hydrogène. Il est urgent de déployer rapidement une stratégie ambitieuse dans ce domaine.

que les Français ont constituée au cours des deux épisodes de confinement ne demande qu'à être réinvestie. La mobilisation de ces capitaux sera également déterminante pour la réussite du plan de relance.

Le second choc, c'est un choc de simplification. Il s'agit de faciliter le désir d'entreprendre, d'investir et de créer dans notre pays. C'est le grand défi qui nous attend désormais : inventer une nouvelle forme de croissance, adaptée aux impératifs écologiques et territoriaux et libérée des freins inutiles. Cette crise doit permettre à notre pays

est nécessaire, mais elle ne peut se faire qu'en accompagnant les plus touchés par la crise, les plus fragilisés. Monsieur le ministre, le gouvernement auquel vous appartenez a mis en place dès le début de la crise des dispositifs exceptionnels de soutien aux entreprises et aux salariés, lesquels continuent aujourd'hui d'être mobilisables.

Tous les champs des politiques publiques sont concernés, tous les acteurs impliqués : collectivités, administrations, particuliers et entreprises. L'objectif est de rebondir le plus rapidement possible dans un contexte de récession. Alors que nous connaissons une croissance de nouveau négative ce trimestre,

Hors plan de relance, le budget du ministère de la transition écologique augmente de 1,3 milliard d'euros afin de répondre à deux objectifs : décarboner notre économie, en réduisant nos émissions de carbone de 40 % d'ici à 2030, et soutenir nos secteurs d'avenir, en misant sur les technologies vertes. Des crédits seront également fléchés vers la filière de la pêche, qui connaît de nombreux bouleversements hors crise sanitaire, vers la lutte contre l'artificialisation des sols, en soutien à l'économie sociale et solidaire et aux circuits courts ; vers le renforcement de notre souveraineté agricole et alimentaire grâce à l'accélération de la transition agroécologique.

sécurise les approvisionnements critiques et la relocalisation de projets industriels. Près de cent trente dossiers, portant sur des investissements supérieurs à 1 million d'euros, ont déjà été déposés dans le cadre d'un appel à projets

faut sécuriser le passage à l'âge adulte, rendu encore plus difficile en cette période chaotique, et à l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés. Pour financer cette relance, le Gouvernement s'appuiera également sur les 40 milliards d'euros de l'Union européenne, obtenus grâce à l'accord de juillet. Saluons l'action résolue et efficace de nos eurodéputés, qui se battent encore contre certaines résistances. Je pense à Valérie Hayer, députée européenne et rapporteure sur les ressources propres de l'Union, qui a été auditionnée la semaine dernière par la commission des affaires européennes. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, les Européens empruntent en commun pour investir ensemble. En plus des crédits, l'articulation des différentes aides et des différents opérateurs est fondamentale, notamment avec les collectivités territoriales. le rôle de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et celui des sous-préfets à la relance est primordial. Au cours des prochains mois, nous devrons rester vigilants

qui souffre particulièrement de la crise pour ses études et l'accès au marché du travail. Nous voterons bien entendu les crédits qui nous sont présentés aujourd'hui. La parole

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs la mission « Plan de relance », avec ses 36,4 milliards d'euros d'autorisations d'engagement et 22 milliards d'euros de crédits de paiement, rassemble une multitude de dispositions relevant habituellement d'autres missions. Elle mélange le court et le moyen terme, le fonctionnement et l'investissement, entretenant ainsi une certaine confusion, source d'un manque de lisibilité.

La construction hétéroclite de ces programmes budgétaires suscite des inquiétudes sur les conditions de leur exécution, car il y a un risque de confusion lors de leur mise en oeuvre.

Comme je l'ai déjà indiqué lors de la discussion générale sur la première partie du projet de loi de finances, je déplore que cette mission ne mobilise pas suffisamment de moyens pour soutenir les collectivités territoriales, pour faire face à la gestion de la crise sanitaire, d'autre part, pour participer à la relance économique. Leur rôle de levier est pourtant prépondérant pour le tissu économique et social de nos territoires. Les associations d'élus du bloc communal s'inquiètent du manque de confiance et de la faiblesse des crédits accordés aux territoires par le Gouvernement. Leurs marges de manoeuvre financières et fiscales ne cessent d'être rognées et les ressources locales s'érodent encore davantage avec la crise sanitaire. sanitaire. Les petits commerces pourront rouvrir ce samedi, mais combien se relèveront de façon pérenne ? Quel avenir se dessine pour le secteur de la restauration et du tourisme et, par voie de conséquence, pour la viticulture ? Ce sont les piliers de l'économie de mon département, l'Hérault. Quel avenir également pour la culture ? Toutes ces questions appellent une réponse politique forte pour soutenir un redémarrage rapide des trains de l'activité, avec les collectivités locales en locomotives. sont des interlocutrices privilégiées qui devraient être associées à la définition des projets, matérialisés par les contrats régionaux ou infrarégionaux de relance, au pilotage des crédits et à leur suivi dans le cadre des comités régionaux et départementaux.

Monsieur le ministre, que sont les 100 milliards d'euros devenus ? Le manque le plus évident de ce plan réside dans l'absence quasi totale de mesures visant à stimuler la demande.

M. Bruno Le Maire, abondamment cité dans cet hémicycle, malheureusement jamais présent pour pouvoir s'en réjouir, déclarait à l'Assemblée nationale en juillet dernier : « La France n'a pas de problème de demande, il n'y a donc pas de plan de relance de la consommation, pas de renforcement des transferts sociaux ni de développement de l'emploi public ». Ce choix a des conséquences très claires d'un point de vue social : les plus fragiles de nos concitoyens n'ont pas grand-chose à attendre de ce plan. Le soutien aux personnes précaires s'établit à 800 millions d'euros, soit 0,8 % du plan, ce qui inclut la revalorisation ponctuelle de l'allocation de rentrée scolaire, le ticket-restaurant à un euro et le soutien à l'hébergement d'urgence.

l'instar de ce qui s'est fait dans notre pays au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La relance ne passera donc pas par la relance de la consommation, notamment pour les plus fragiles. Bien au contraire,

Le coeur de ce plan n'a donc rien à voir avec la relance. C'est d'abord la reprise de la politique de l'offre du Gouvernement Philippe qui est accélérée, avec une baisse massive des impôts de production pour 20 milliards d'euros sur deux ans. Pour le Gouvernement, ces baisses devraient permettre de réindustrialiser la France, mais il ne demande aucune garantie à cet égard. S'agissant des grands groupes, nul ne sait si cet argent ne finira pas à terme en dividendes, en épargne personnelle, en investissements à l'étranger ou sur les marchés financiers. valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va d'abord profiter aux plus grandes entreprises. Selon de nombreux économistes, un quart de cette baisse profitera à 280 entreprises, tandis que 250 000 autres, les plus petites, n'y gagneront que 125 euros. L'aspect massif de ce plan cache en réalité une diffusion lente propre à la politique de l'offre. Sur les 100 milliards d'euros claironnés, seulement 30 milliards seront disponibles l'an prochain. Nous sommes très loin du des années 1930. Nous pensons que ce plan de relance est largement sous-calibré face à la crise que nous traversons. Le Gouvernement prévoit qu'il permette d'augmenter la croissance de 1,5 point en 2021

sans catastrophisme. Le débat sur la dette est un débat politique. Magritte a peint un tableau célèbre, en 1928, accompagné de la légende : « » Monsieur le ministre, ceci n'est pas un plan de relance

après le plan d'urgence, après le plan de soutien, après les adaptations successives de l'un, puis de l'autre, l'heure est enfin venue d'examiner les crédits alloués au plan de relance. En responsabilité, suivant notre rapporteur spécial, je vous le dis sans attendre, monsieur le ministre, nous soutiendrons ce plan de relance ; mais, au fond de nous, il y a beaucoup de regret devant le temps perdu. Alors que le PIB dégringolait de près de 14 points au deuxième trimestre 2020 et que nos voisins européens dégainaient différentes mesures favorables à la relance de leur économie, la France a, elle, attendu fin septembre pour présenter les siennes. Dès l'été, le Sénat avait pourtant alerté le Gouvernement sur la nécessité d'une réponse rapide afin d'endiguer les difficultés sociales et de limiter autant que possible les défaillances en cascade de nos entreprises. Le chiffre rond de 100 milliards d'euros est martelé avec beaucoup de conviction. Mais, à y regarder de plus près, la réalité de ce plan de relance est beaucoup plus ambiguë qu'il n'y paraît, car l'enveloppe globale est artificiellement gonflée. Vous conjuguez des crédits déjà « budgétés » en 2020 avec d'autres qui ne le seront, au mieux, qu'en 2022. Vous agrégez des mesures tantôt budgétaires, tantôt fiscales, tantôt conjoncturelles, tantôt structurelles ; des sources de financement tantôt nationales, tantôt européennes, tantôt certaines, tantôt hypothétiques. Nous aimerions à cet égard avoir quelques précisions sur la traduction concrète du plan de relance européen à l'échelle du pays. Vous créez une mission, mais mobilisez en dehors plus de 15 milliards d'euros d'autorisations d'engagement. Comment s'y retrouver ? Au bout du compte, seuls 22 milliards d'euros de crédits de paiement seront consacrés l'année prochaine au plan de relance, soit 1 % seulement de la richesse nationale ... Préjudiciable pour la confiance des acteurs de terrain, qu'ils soient économiques ou politiques, le manque de clarté l'est finalement aussi pour l'efficacité de la gestion des aides attribuées. En confiant les manettes à Bercy, autrement dit à l'État central, vous prenez le risque d'entraver le déploiement effectif de la relance dans les territoires. Là aussi, nous avons lancé l'alerte depuis plusieurs mois mois : la réussite de la reprise économique ne pourra s'obtenir qu'en concertation avec les collectivités locales et leurs élus. Un mot enfin sur le volet social de ce plan de relance. Le mécanisme d'activité partielle a formé un filet de sécurité bienvenu pour bon nombre de salariés. Nous accueillons aussi favorablement le dispositif d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Des trous dans la raquette demeurent toutefois, concernant tout à la fois les travailleurs indépendants, les intérimaires, les emplois précaires et les chômeurs. Les crispations sociales appellent également un devoir d'exemplarité. C'est pourquoi nous soumettrons à l'approbation de la Haute Assemblée un amendement visant à contrecarrer l'effet d'aubaine créé par l'allocation de fonds au profit de grandes entreprises qui seraient tentées par les délocalisations. Pour l'engagement des mesures d'urgence et l'extension des mesures de soutien, le groupe Union Centriste a fait son devoir, et il va encore le faire aujourd'hui avec l'adoption des crédits de la mission. monsieur le ministre, nous vous le disons avec la franchise qu'autorise le débat parlementaire, notre soutien aujourd'hui ne sera pas sans exigences pour l'avenir. La parole

100 milliards d'euros. Après analyse, on trouve de tout, cela a été dit : des mesures déjà engagées en 2020, pour 15 milliards ; la baisse des impôts de production, une vieille lune, pour 20 milliards ; le financement du Ségur de la santé, des participations d'organismes variés qui, pour l'essentiel, ne font qu'accélérer leurs programmes, et 49 milliards de crédits budgétaires, dont 36 milliards au strict titre de cette mission et 22 milliards en crédits de paiement.

Ces discours grandiloquents lassent ou inquiètent. On ne fait qu'inquiéter les Français, qui se disent que demain il faudra rembourser et qui, du coup, économisent au lieu de consommer. Si c'est l'objectif recherché, alors c'est réussi Finalement, pourquoi une mission spécifique ? Sans doute pour mieux séparer des charges temporaires des dépenses ayant vocation à devenir récurrentes. On pourrait sans doute s'interroger sur la conformité de cette présentation à la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, tant certaines dépenses auraient pu trouver tout naturellement leur place dans les missions budgétaires. Malheureusement, la baisse des impôts de production, elle, est présentée comme ayant vocation à être pérenne. Au-delà du fait que le lien avec la relance économique reste à démontrer, comment peut-on aujourd'hui proposer une réforme visant à priver l'État de 10 milliards d'euros par an au moment où la dette explose ?

En témoignent les timides avancées vers une taxation exceptionnelle des suppléments de recettes des assurances ou des géants de l'e-commerce. Rémi Féraud reviendra sur les priorités de notre groupe qui semblent manquer dans votre plan de relance. Je voudrais pour ma part évoquer la situation des jeunes dans notre pays. Quelques constats : en 2018, le taux des 18-29 ans vivant sous le seuil de pauvreté s'élevait à 12,5 %, soit 4,2 points de plus que la moyenne nationale. Les jeunes sont les premières victimes des chocs économiques. Les effets de la crise sanitaire ont été immédiats, puisque le chômage des jeunes a bondi de 2,6 points sur un an au troisième trimestre 2020, contre 0,6 point pour la moyenne nationale. Le plan « un jeune, une solution » n'apporte à ce problème qu'une réponse lacunaire, puisqu'au jeune qui ne parviendrait pas à s'inscrire dans l'un des parcours d'insertion, la « solution » proposée se limiterait aux aides ponctuelles de solidarité, comme celles versées à l'été et à l'automne 2020. Je constate d'ailleurs que la ministre du travail est revenue en partie sur ce point ce matin. Si l'on peut noter un renforcement bienvenu des différents dispositifs de la politique de l'emploi, force est de constater que rien ne garantit que les instruments mis en place bénéficient prioritairement aux jeunes les plus en difficulté. Surtout, ce plan revêt un caractère strictement conjoncturel, alors même que le problème de la pauvreté des jeunes, s'il est accentué par la crise, est bel et bien structurel. Ceux-ci seraient d'ailleurs fortement affectés par la décision obstinée du Gouvernement de maintenir la réforme de l'assurance chômage. En rendant plus restrictives les conditions d'ouverture des droits pour les personnes ayant alterné périodes de chômage et contrats courts, cette réforme pénaliserait avant tout les jeunes, comme l'a démontré l'Observatoire des inégalités. Aujourd'hui, les conditions d'accès des jeunes aux minima sociaux sont particulièrement limitées, notamment aux jeunes parents et à ceux ayant travaillé au moins deux ans à temps plein au cours des trois dernières années. Près d'un million de jeunes peuvent certes bénéficier d'aides au logement, mais celles-ci ne sauraient être assimilées à un revenu d'existence. La garantie jeunes constitue un dispositif important d'accompagnement vers l'autonomie des jeunes les plus éloignés du marché de l'emploi, mais, avec une éligibilité limitée à dix-huit mois, elle ne saurait apporter de réponse globale au problème de la pauvreté des jeunes. La France est l'un des rares pays européens dans lesquels les minima sociaux ne sont pas accessibles aux jeunes de moins de 25 ans. À cet égard, je vous renvoie au rapport de Christophe Sirugue en 2016. L'épreuve de la crise doit constituer pour nous l'occasion de reconstruire un lien de confiance entre les générations, en pensant collectivement un nouveau cadre pour favoriser l'émancipation des jeunes adultes. C'est la raison pour laquelle le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de financer en 2021 le lancement d'une expérimentation territoriale visant à instaurer une dotation une dotation d'autonomie pour la jeunesse, permettant d'apporter un soutien monétaire aux jeunes émancipés. Monsieur le ministre, le soutien aux entreprises comme aux salariés et aux indépendants est fondamental. Celui que nous devons aux plus fragiles et à notre jeunesse, cette jeunesse qui demain, avec nous, devra gérer la dette creusée par cette pandémie, l'est tout autant. Ce plan de relance ne le dit que trop peu.

Lavarde. La pandémie de covid-19 et ses conséquences sur notre économie justifient aujourd'hui l'interventionnisme de l'État. Le chiffre de 100 milliards d'euros, sur lequel le Gouvernement communique largement, est impressionnant ; c'est quatre fois plus qu'après la crise de 2008. Il se pourrait pourtant que les montants ne soient pas réellement décaissés. En juillet, le Président de la République s'est réjoui de l'accord du Conseil sur le plan de relance européen, mais je voudrais tempérer quelque peu cet enthousiasme. En effet, les 40 milliards d'euros qui devraient être alloués à la France sont soumis à un certain nombre de contreparties. Notamment, la France va devoir présenter son plan à la Commission au début de l'année prochaine. Dès mercredi 18 novembre dernier, la Commission s'est inquiétée de la conséquence de la baisse des impôts de production sur la soutenabilité de notre dette à moyen terme. Pourtant, les analyses économiques sont assez unanimes pour dire que la baisse des impôts de production est la mesure de ce plan de relance qui aura le plus d'effet sur la croissance de moyen terme. Il se pourrait donc, parce que nous n'allons pas respecter les critères de conditionnalité, qu'une partie des aides de l'Union européenne ne nous soit jamais allouée. Au-delà du débat sur le montant réel du plan, je formulerai trois critiques sur son contenu. Tout d'abord, il me semble que ce plan procède un peu de l'économie circulaire : des idées plusieurs fois évoquées reviennent sans que soient apportées de véritables réponses à des faiblesses déjà identifiées.

Un focus est opéré sur le fret ferroviaire, avec la gratuité des péages ou des mesures en faveur du wagon isolé. Mais, quelle est l'articulation avec les travaux de régénération ? Avec quels sillons ? Ce sera le quatrième plan fret en vingt 6,7 milliards d'euros sont fléchés vers la rénovation thermique des bâtiments. Le « grand plan d'investissement » de l'automne 2017 accordait déjà 9 milliards d'euros à cette politique que nous soutenons, au regard du poids du logement dans notre bilan carbone. Cependant, une étude de l'École des mines de 2019 révèle que le taux de rentabilité de la politique de rénovation thermique sur le seul critère des économies d'énergie est de cent vingt ans ! Si l'on s'en tient aux résultats de cette étude, il faudrait plutôt concentrer concentrer les moyens publics vers les fournisseurs, de manière à ce qu'ils améliorent la qualité de la rénovation et qu'ils en diminuent le coût, plutôt que vers les consommateurs. C'est d'autant plus indispensable, si l'on veut engager ce mouvement dans la durée, que le budget de MaPrimeRénov'n'est augmenté que temporairement. 1,2 milliard d'euros sont fléchés vers l'agriculture : souveraineté alimentaire, transition agroécologique, accompagnement de l'agriculture et de la forêt dans l'adaptation au changement climatique Des thèmes qui ne sont pas nouveaux. Mais quelles sont les réponses aux problèmes structurels de notre agriculture ? La ferme France perd de la valeur ajoutée, de l'emploi et de la compétitivité. Le Président de la République, lors de la présentation du plan de relance, a dit : « La véritable ambition de France Relance n'est pas tant dans l'importance des moyens mobilisés pour soutenir l'activité à court terme, que dans la philosophie de transformation qui sous-tend le plan. » » Or cette transformation ne transparaît pas dans le saupoudrage qui nous est proposé : 38 mesures ont un coût inférieur à 1 milliard d'euros. Le caractère très divers des mesures rend difficile l'appréciation du plan sur l'économie. Je cite pêle-mêle : modernisation des centres de tri, plantation de 7 000 kilomètres de haies, soutien à l'accueil des animaux abandonnés, développement de jardins partagés, réseau radio haut débit, acquisition de caméras piétons ... Et en même temps : développement de la filière de l'hydrogène vert, soutien au nucléaire et à l'aérospatiale. Quelle est donc votre véritable vision de l'économie française dans dix ans ? Il n'y en a pas ! Je l'ai déjà dit, nous pensons que ce plan est trop tardif. Seuls 25 milliards d'euros seront consommés fin 2021 la totalité de l'enveloppe ne le sera qu'en 2025. Dans le même temps, la quasi-totalité du plan de relance de l'Allemagne devrait être déployée d'ici à la fin de l'exercice 2021. Nous sommes aussi un peu inquiets quant à la mise en oeuvre. Le 30 août, la ministre de la transformation et de la fonction publiques indiquait que les sous-préfets à la transformation et à la relance auraient pour mission de faire « remonter tous les blocages administratifs de procédures, de dispositifs très compliqués Ce plan de relance est un pari pour relancer l'économie ; c'est un pari sur l'offre. Nous croyons à cette option, car c'est la seule à même de développer la croissance potentielle de l'économie française et ainsi d'avoir un effet à long terme sur l'emploi. Mais c'est aussi un pari sur notre capacité à engager des réformes structurelles pour dégager des excédents permettant de rembourser la dette covid. C'est un véritable pari qui engage les gouvernements sur plusieurs quinquennats. En effet, l'emprunt commun européen ne commencera à être remboursé qu'en 2028, sur la base de conditions qui ne sont pas encore connues.

Estrosi Sassone. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le plan de relance consacre environ 7 milliards d'euros au secteur du bâtiment ; ce chiffre impressionne. À l'échelle des 100 milliards du plan de relance, la part qui lui est dévolue correspond en fait à son poids dans l'économie nationale. Si l'on pousse l'analyse, plusieurs questions se posent : la rénovation thermique bénéficie de moyens supplémentaires, mais sont-ils à la hauteur ? La construction neuve n'a-t-elle pas été oubliée ? Quant aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, les maires qui ont signé l'appel du 14 novembre dernier nous disent combien le compte n'y est pas. La rénovation thermique des bâtiments, tout d'abord, est bien la principale destinataire des crédits, avec une enveloppe d'environ 6,7 milliards 4 milliards sont attribués aux bâtiments publics, 200 millions aux locaux des TPE-PME et 500 millions aux bailleurs sociaux. En outre, 2 milliards d'euros seront attribués aux particuliers dans le cadre de MaPrimeRénov'. Cette prime réintégrera tous les Français, bailleurs comme locataires ; surtout, elle s'ouvre aux copropriétés, ce qui est une bonne chose. Deux bémols subsistent toutefois. Le premier, c'est que, loin de correspondre à des crédits nouveaux, MaPrimeRénov'recycle très largement les moyens précédemment dévolus au crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, qui dépassaient 1,1 milliard d'euros par an. De ce fait, on se demande comment cet élan se poursuivra après le plan de relance, c'est-à-dire après 2022. Le second bémol, c'est le grand décalage entre les moyens déployés- 2 milliards d'euros -et le chiffrage de la transformation des logements évoqué par la Convention citoyenne pour le climat, qui s'élève à plus de 20 milliards, soit dix fois plus.

Aussi étonnant que cela puisse paraître : rien ! Elle est dans l'angle mort du plan de relance. Pourtant, la situation est grave. Malgré le rebond observé après le premier confinement, les professionnels estiment que l'on devrait atteindre moins de 350 000 permis de construire. Au total, sur 2020-2021, on déplorera sans doute 100 000 constructions de logements de moins. J'avais déjà averti à cette tribune : après la crise sanitaire arrive la crise du logement. Face à cette situation, les solutions mises en oeuvre par le Gouvernement sont insuffisantes, alors que l'on considère que 100 000 logements construits équivalent à 200 000 emplois préservés ou créés. Le secteur du bâtiment a arraché la prolongation des dispositifs d'investissement locatif intermédiaire Pinel et d'aide à l'accession sociale au travers du prêt à taux zéro, le PTZ, mais ce ne sont pas là des mesures nouvelles. Ce n'est pas une relance. D'autres mesures étaient possibles, comme le retour à une TVA de 5,5 %, au lieu de 10 %, pour les logements sociaux. Ce taux réduit représente 5 000 euros de moins par logement. On comprend l'effet massif que l'on peut obtenir, en l'appliquant à plusieurs dizaines de milliers de logements par an. On pouvait également soutenir les opérations de reconversion de locaux en logements ou encore l'accession à la propriété au travers du rétablissement de l'APL-accession, injustement supprimée il y a deux ans. On pouvait également prendre des mesures structurelles, en libérant les bailleurs sociaux du poids de la réduction de loyer de solidarité, la RLS, qui pèse 1,3 milliard d'euros par an, ou créer enfin un véritable statut du bailleur privé, qui ne doit plus être considéré comme un rentier improductif, mais bien comme un entrepreneur en logement. Enfin, les quartiers populaires sont les oubliés de ce plan de relance. Trois ans après le discours de Tourcoing, le constat est amer. Le rapport Borloo est resté lettre morte. Ces quartiers sont aujourd'hui en plein désarroi. Partout, sur le terrain, les signaux sont au rouge. Les quartiers populaires sont deux fois plus infectés par la covid-19 en raison de l'exiguïté des logements. De plus, la crise sanitaire a provoqué une très grave crise économique et sociale. Les maires de ces quartiers dénoncent aujourd'hui une véritable non-assistance à des territoires en danger de décrochage de la République.

de 10 millions d'euros cette année. En 2008, au contraire, des mesures spécifiques importantes et rapides avaient été prises pour les quartiers par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ces maires demandent 1 % du plan de relance : alors, écoutez-les, monsieur le ministre, pour résorber cette fracture territoriale

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débutons l'examen des crédits de la mission « Plan de relance » et j'aimerais m'arrêter sur plusieurs points chers à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable que j'ai l'honneur de présider. Mon premier point est un motif de satisfaction. La nouvelle mission consacre 240 millions d'euros au déploiement de la fibre dans le cadre du plan France Très haut débit. Ces crédits s'ajoutent aux 30 millions d'euros ouverts par la troisième loi de finances rectificative, à l'initiative de notre assemblée, et aux 280 millions de crédits « recyclés » promis par le Gouvernement en début d'année. En cumulé, avec 550 millions d'euros, les moyens pourraient être suffisants pour un déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire d'ici à 2025.

J'ai un second motif de satisfaction sur ce plan de relance concernant les efforts budgétaires consentis en faveur de la sécurité des ponts. La mission d'information conduite par notre commission l'année dernière avait dressé un constat un constat alarmant sur ce sujet et mis en évidence le fait que de nombreux ponts gérés par les collectivités territoriales sont en mauvais état. Nous avions recommandé la mise en place d'un « plan Marshall » et la création d'un fonds d'aide aux collectivités territoriales doté de 130 millions d'euros par an. Les crédits prévus par le plan de relance constituent donc une première étape importante qui permettra d'aider les collectivités à recenser et à diagnostiquer l'état de leurs ponts. elle reste insuffisante ; il faut aller plus loin et aider les petites collectivités qui n'ont pas les ressources suffisantes pour réparer leurs ponts en mauvais état. Tel est le sens d'un amendement qui sera présenté tout à l'heure au nom de la commission. Enfin, s'agissant de la prévention des risques et de la lutte contre les pollutions de toutes natures, je salue le renforcement des moyens de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Ademe. Ces différents motifs de satisfaction n'empêchent pas pour autant quelques inquiétudes. Je regrette en effet le manque d'envergure du plan de relance sur la question des risques naturels, alors que, vous le savez, un euro investi dans la prévention permet d'économiser à terme sept euros de travaux. Sur le secteur ferroviaire, je regrette que le plan de relance n'aille pas plus loin. Les moyens consacrés à la régénération du réseau et à la remise en état des petites lignes restent inférieurs aux préconisations du rapport Philizot. Quant au fret, les mesures sont évidemment bienvenues, mais cette première étape devra être intensifiée

une part importante des montants prévus recouvre soit la compensation de pertes et de retards liés à la crise, soit des dépenses déjà prévues, mais non budgétées. Enfin, ce manque d'ambition se constate également en matière de protection de la biodiversité. Les moyens ne sont pas à la hauteur de nos ambitions face aux récentes et constantes alertes sur l'état de la biodiversité, sans rappeler son lien avec la crise sanitaire actuelle. La parole

les crédits inscrits dans ce plan de relance que ceux qui n'y sont pas, c'est-à-dire le plan d'urgence dont notre pays a besoin dans la crise et qui manque cruellement. Ce plan gouvernemental a le mérite d'exister, mais il n'est pas si grand que la communication qui l'accompagne, et surtout il est incomplet : c'est pourquoi nous avons présenté un budget alternatif, dont les mesures seront illustrées par nos amendements. Car comment oublier les jeunes, cette génération sacrifiée à la fois par la crise sanitaire et ses répercussions économiques ? Parce qu'il n'est pas normal que notre pays laisse tant de jeunes tomber dans la pauvreté, nous proposerons la création d'une dotation d'autonomie pour destinée aux 18-25 ans, leur permettant de disposer des ressources auxquelles ils n'ont plus accès en raison des restrictions actuelles d'activité. Et parce que chaque jeune porteur d'un projet associatif ou professionnel doit pouvoir se faire aider, particulièrement dans cette période, nous proposerons aussi de renforcer le financement de ces projets. Face à la crise que nous traversons, il est évidemment impératif de relancer l'activité économique, mais il n'est pas possible pour autant de faire abstraction du défi climatique. C'est pourquoi nous devons accélérer dans le développement d'offres de transports propres, tant en milieu urbain que dans les zones rurales. Nous proposerons, dans ce sens, un « choc écologique » des transports, en plus d'un soutien spécifique destiné aux territoires ruraux. nous l'avons déjà fait remarquer au cours de nos débats, ce projet de loi fait la part belle aux grandes entreprises. Toutefois, parce que la transition écologique ne passera pas seulement par les multinationales, nous voulons créer un fonds de transition écologique destiné exclusivement aux TPE et aux PME. Vous le voyez, nous n'opposons pas le développement économique et la transition écologique, non plus que le développement économique et la justice sociale. À la politique de l'offre du Gouvernement, nous ajoutons

Pour soutenir le monde associatif et le secteur culturel si touchés par cette crise, nous proposons aussi un total de 800 millions d'euros répartis en un plan de soutien à la vie associative et un renforcement des aides à la culture.

Le Ségur de la santé ne doit être qu'un premier pas. Nous voulons un grand plan pour l'hôpital et l'autonomie. Notre pays, mes chers collègues, a besoin d'un choc social et écologique

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les présidents

Les 86 milliards d'euros restants seront financés par l'État. Il s'agit de 20 milliards d'euros sur deux ans de baisse des impôts de production. Cette baisse bénéficiera- je le précise -à 542 000 petites et moyennes entreprises et à 25 000 entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises.

en complément des 10 milliards d'euros dont le décaissement est prévu dès l'année 2020. Le reste des crédits de paiement sera ouvert pour les années 2022 et suivantes. La mission comporte trois programmes budgétaires qui reprennent les priorités du plan de relance. Nous avons souhaité que cette mission, massive- elle représente, je le rappelle, plus de 36 milliards d'euros -, ne soit divisée qu'en trois programmes afin de garantir la plus grande fongibilité, de pouvoir le cas échéant faire jouer la clause de revoyure et de nous assurer de la mise en oeuvre de la totalité du plan de relance avec le plus de souplesse possible. certains, au vu de la situation sanitaire, le montant de l'investissement devrait être actualisé et il faudrait l'augmenter. Je ne suis pas de cet avis. Les 20 milliards d'euros supplémentaires votés en PLFR 4 pour renforcer les mesures d'urgence permettront à l'économie française de se trouver, une fois les incertitudes sanitaires levées,

d'une attribution automatique au vu de la délivrance des permis de construire et des projets. La relance est donc d'ores et déjà à l'oeuvre partout en France ; la grande majorité des investissements prévus sera réalisée dans les deux prochaines années.

Elle sera évidemment totalement décaissée dans les meilleurs délais, puisque l'ensemble des projets sera annoncé d'ici à la fin du mois de novembre. Nous aurons à tenir avec Bruno Le Maire une conférence de l'immobilier public de l'État et des universités pour déterminer la liste des projets soutenus.

Sans les territoires, elle serait désincarnée ; elle ne serait pas concrète. Pour retrouver notre confiance collective, la relance doit se voir partout, dans les quartiers prioritaires, dans les bourgs ruraux, dans les zones d'activités ou dans les foyers.

régionalisés. Troisièmement, il y a des mesures dont les paramètres sont définis au niveau ministériel, mais dont la gestion sera déconcentrée, car les préfets et les services déconcentrés sont les plus aptes à identifier pour chaque thématique les projets pertinents sur les territoires. seront déconcentrés au fur et à mesure de la réalisation des projets locaux, pour garder si nécessaire une faculté de redéploiement entre les différentes mesures du plan. Une attention particulière sera portée aux investissements ayant des résultats immédiats pour les Français, notamment dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des déchets.

La contractualisation avec les collectivités dans le cadre du déploiement du plan de relance sera pragmatique. Elle sera effectuée avec les collectivités qui le souhaitent. Elle n'aura pas d'autre objectif que la formalisation du cofinancement afin de favoriser la rapidité de l'exécution. Elle permettra d'associer les collectivités au financement des projets pour créer un effet de levier sur les crédits de l'État. L'accord de méthode signé entre l'État et les régions consacre ainsi la place de ces dernières au sein du plan de relance, en prévoyant notamment que les montants investis par elles dans les contrats de plan conclus avec l'État pour la période 2021-2027 ne sauraient être inférieurs à 20 milliards d'euros. De son côté, l'État inscrira dans des accords régionaux de relance les dépenses du plan, qui seront réalisées seulement sur un territoire donné. l'échelon infrarégional, les collectivités pourront aussi souscrire le contrat de relance pour 2020-2026. Les instructions nécessaires à leur mise en oeuvre ont été adressées aux services déconcentrés.

Ainsi que l'a annoncé le Président de la République mardi soir, nous allons continuer à les soutenir aussi longtemps que la crise durera. Nous allons renforcer les aides apportées aux secteurs qui ne pourront rouvrir au plus tôt que le 20 janvier : les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques.

prolongation des périodes d'exonération de cotisations ou l'activité partielle sur les premiers mois de l'année, au bénéfice des secteurs les plus touchés par la crise ou de ceux qui verront leur activité durablement entravée par les mesures administratives. Le montant des crédits sera proposé au Parlement en nouvelle lecture du projet de loi de finances. Un certain nombre d'estimations ont été rendues publiques. Vous avez évoqué les chiffres qui ont été rapportés par la presse sur le coût des nouvelles options que nous envisageons. Je pense notamment à la prise en charge

la reprise de l'activité sera progressive, que nous n'aurons pas à vivre un troisième confinement et que les mesures administratives seront progressivement allégées. Cela nous oblige à un calcul plus fin de l'estimation du coût, mois par mois, sur une pente que nous souhaitons évidemment dégressive. Ce travail est en cours de finalisation.

des crédits dans le PLF. Je veux terminer, en nous invitant collectivement à la confiance et en rappelant à la fois les défis que nous avons à relever ensemble et les succès que nous connaissions voilà un peu moins d'un an, à la fin de l'année 2019. La croissance était solide. Le chômage était passé sous les 8 % dans l'Hexagone. Les levées de fonds en capital-risque étaient en expansion. La France était devenue le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Le troisième trimestre de cette année constitue un autre motif d'espoir. Dès la sortie du confinement, notre économie a connu le rebond le plus fort de tous les pays d'Europe, avec 18,2 % de croissance au troisième trimestre. signe de sa résistance, de sa capacité à repartir et de la confiance des acteurs économiques. Au-delà de l'appréciation des uns et des autres sur le plan de relance,

le chômage. Je crois, et vous êtes nombreux à y croire également, à la capacité de notre économie à retrouver les succès que nous connaissions précédemment. Je crois aussi à un sursaut collectif. Je suis convaincu- je sais que ce n'est pas partagé par tous -que nous traversons cette crise de la meilleure des manières possible, en n'augmentant pas les impôts et n'en créant pas de nouveau. Nous continuerons à investir dans les secteurs clés pour notre prospérité et notre souveraineté. Je pense à l'hydrogène, qui a été cité, aux batteries électriques, aux technologies quantiques, à l'intelligence artificielle. Nous continuerons à simplifier la vie quotidienne des entreprises, des Français, des usagers, des contribuables. Je pense à la contemporanéisation du crédit d'impôt pour les services à la personne dans quelques mois, à l'unification du recouvrement, à la création d'outils uniques de recouvrement des créances fiscales et sociales des entreprises et des particuliers. Nous continuerons à valoriser l'emploi, à protéger les compétences, en particulier dans le cadre de l'activité partielle de longue durée. Nous continuerons à travailler à la compétitivité, à l'innovation et à la formation, comme nous nous sommes engagés à le faire depuis le début du quinquennat.

Notre volonté est que ce plan de relance soit totalement dédié à la reprise, à la relance et au soutien de notre économie, avec une garantie : l'efficacité de ce plan de relance, qui nous permettra de tourner la page de la crise et de ses conséquences économiques et sociales. Nous allons

qui vise à assurer le financement du plan de prévention du risque sismique au bénéfice des hôpitaux des Antilles, à hauteur de 10 millions d'euros par an pendant trois ans. Intégré au Ségur de la santé, ce financement sera assuré par l'assurance maladie, puis par l'agence

Cet amendement tend ainsi à annuler les crédits ouverts à ce titre sur la mission « Plan de relance » à hauteur de 30 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 10 millions d'euros en crédits de paiement.

Cet amendement est dans la lignée de l'une de leurs propositions : développer un plan d'investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares afin d'en faire des pôles multimodaux. Un tel plan d'investissement dans le secteur du ferroviaire est un levier central pour hâter la décarbonation des transports, qui sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre en France, à hauteur de 30 %. Le ferroviaire, lui, ne représente que 0,3 % des émissions de CO2 de l'ensemble du secteur des transports, alors qu'il transporte 11 % des passagers et 9 % des marchandises. Son développement sera donc déterminant sur le front climatique. Il faut donc abonder le ferroviaire. Monsieur le ministre, votre plan de relance ressemble davantage à un plan de soutien à SNCF Réseau pour permettre de préserver l'existant. Il ne pourra guère soutenir la trajectoire bas-carbone. Le plan gouvernemental de 4,75 milliards d'euros étalés sur deux ans couvre en réalité 4,1 milliards d'euros pour préserver les capacités d'investissement de SNCF Réseau et maintenir les travaux de régénération déjà engagés. 650 millions d'euros constituent de nouveaux crédits d'investissement spécifiquement dédiés aux petites lignes, au fret ferroviaire et aux trains de nuit. Avec seulement 14 % du montant du plan dévolu aux nouveaux crédits d'investissement, peut-on parler de plan de relance du ferroviaire ? vise donc à engager un véritable plan, en investissant 3 milliards d'euros supplémentaires par an dans la régénération et la modernisation du réseau ferré et le renouvellement du matériel roulant.

Alors que le Gouvernement refuse tout geste en faveur des plus précaires, l'aggravation de la crise sociale consécutive au deuxième confinement rend ce refus intenable.

C'est pourquoi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat propose la mise en place d'une dotation d'autonomie pour la jeunesse. Il est aujourd'hui primordial d'éviter le creusement sans précédent des inégalités qui frappent une jeunesse mise à très rude épreuve par la crise. Cet amendement n'a pas d'autre objet que de préserver l'égalité des chances pour toute une jeunesse qui porte l'activité de demain, donc l'avenir de notre société.

l'avis du Gouvernement ?

Le Gouvernement l'affirme avec raison, les transports et les mobilités de demain sont un levier indispensable de la relance pour accélérer la transition écologique de notre pays. On peut se réjouir que 11,5 milliards d'euros aient été dédiés aux transports en 2020 et 2021,

1,2 milliard d'euros pour les mobilités du quotidien, dont 700 millions d'euros pour les transports en commun d'Île-de-France et 330 millions d'euros pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) du reste de la France.

Nous nous retrouvons ainsi avec 330 millions d'euros, même pas l'équivalent de deux stations de métro, à partager entre les 337 AOM que compte notre pays, soit 1 million d'euros par AOM. On est bien loin de la relance par l'investissement proclamée par le Gouvernement

écologique absolu, alors que notre pays est pointé du doigt par ses partenaires européens pour le non-respect systématique des règles européennes en matière de pollution aux particules fines et que cette pollution provoque entre 48 000 et 76 000 décès prématurés par an.

C'est un impératif économique, territorial et écologique. Quel

Cet amendement, qui prolonge nos propositions pour que le plan d'urgence soit à la hauteur de la situation sociale que nous constatons toutes et tous sur le terrain,

un récent rapport du Secours catholique estime que la pauvreté touchera à la fin de l'année 2020 près de 10 millions de nos concitoyens. Le plan France Relance que vous défendez, monsieur le ministre, dédie une part importante des fonds au monde économique.

pour nos concitoyens les plus en difficulté, l'horizon s'obscurcit de jour en jour. J'en veux pour preuve le traitement coercitif que vous faites de la question sociale, comme chacun d'entre nous a pu le constater dernièrement. Il est grand temps que le Gouvernement prenne toute la mesure de la situation. On estime à 2 millions le nombre de bénéficiaires du RSA à la fin de l'année 2020, en hausse de 8 % par rapport à 2019.

Cette proposition a un double mérite : redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens allocataires, mais aussi, et surtout, lutter contre la précarité grandissante qui touche nos concitoyens les plus démunis.

Le plan de relance prévoit déjà 3,6 milliards d'euros en faveur des infrastructures et des mobilités vertes, qui s'ajoutent aux 4 milliards la recapitalisation de la SNCF. Je suis d'assez près ces dossiers et je ne me laisse pas plus que vous, mon cher collègue, enivrer par les chiffres ou abattre par les difficultés.

et en outre-mer ». Ce programme temporaire a vocation à soutenir les entreprises présentes en Corse et outre-mer ayant subi une perte d'exploitation du fait de la crise sanitaire. Ce dispositif bénéficiera aux entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions d'euros assurées pour la perte d'exploitation, mais qui ne peuvent pas faire jouer ce mécanisme assurantiel à cause du vide juridique dont font l'objet les catastrophes sanitaires. Cette prise en charge serait garantie à hauteur de 50 % des pertes d'exploitation. Pour rappel, le confinement a entraîné une baisse d'activité de 35 % en Corse et les outre-mer ont connu, en moyenne, une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 12 millions d'euros par jour de confinement.

de compenser les pertes fiscales recensées dans les documents budgétaires et affectées directement ou indirectement à des organismes culturels. Ensuite, il s'agit de compenser

parole est à Mme Isabelle Briquet. En octobre 2019, les groupes socialistes de l'Assemblée nationale et du Sénat avaient présenté un plan d'urgence pour l'hôpital et l'autonomie. Le Gouvernement et la majorité sénatoriale l'avaient tous deux rejeté, malgré un chiffrage budgétaire cohérent et soutenable. La crise sanitaire que le monde traverse depuis plusieurs mois rend cette proposition encore plus impérieuse qu'elle ne l'était à l'époque : le refus du Gouvernement est à la fois incompréhensible et dangereux. Avec cet amendement, nous proposons un effort financier pluriannuel d'investissement.

le personnel soignant, dont les conditions de travail sont rappelées à chaque journal télévisé. Il est temps de démontrer que l'hôpital est notre bien commun : nous y contribuons avec

Fondé sur les analyses et recommandations du réseau Action Climat, cet amendement a pour objet d'accroître les investissements en faveur des petites lignes pour les porter à 600 millions d'euros par an à partir de 2021.

À une gestion très centralisée, les auteurs du présent amendement veulent opposer la création de dynamiques territoriales reposant sur des stratégies de développement local et sur des coconstructions avec l'ensemble des acteurs présents

de permettre l'amélioration de la vie dans nos territoires, mais aussi de tirer pleinement parti de leur potentiel de développement. En effet, les espaces ruraux disposent de ressources naturelles-

qui sont confrontées à une baisse de leurs recettes et au maintien de certains frais fixes, ces derniers représentant bien souvent une part prépondérante de leur budget. Les associations et structures d'aide alimentaire sont doublement touchées par la crise, dans la mesure où leur public « cible » s'est particulièrement élargi ces derniers mois. La pauvreté et les difficultés à s'alimenter progressent tragiquement dans notre pays. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'apporter une réponse à ces questions. Les associations concernées estiment avoir besoin d'un milliard d'euros d'aides publiques pour répondre aux demandes, auxquelles elles font face sur le terrain au quotidien. de l'importance de ces tissus associatifs locaux, les auteurs du présent amendement estiment qu'il est nécessaire de créer un fonds de soutien au tissu associatif. Ce fonds, qui pourrait être géré de manière territorialisée par le représentant de l'État, aurait vocation à permettre aux structures en difficulté de survivre à la crise que

La rénovation énergétique des bâtiments est une nécessité absolue pour plusieurs raisons : la seule énergie absolument propre est celle que nous ne consommons pas ; l'ensemble des bâtiments résidentiels consomme 44 % de l'énergie en France et émet 123 millions de tonnes de gaz carbonique la diminution de la consommation énergétique permet de faire baisser les factures des ménages, notamment des plus modestes ; la rénovation thermique n'a pas seulement des avantages en termes d'énergie, elle apporte aussi un meilleur confort et permet de réduire la pollution de l'air intérieur et ses effets néfastes sur la santé ; les travaux de rénovation génèrent des centaines de milliers d'emplois.

Pour ces seules passoires énergétiques, l'initiative Rénovons ! estime que les besoins d'investissement s'élèveraient à 3,2 milliards d'euros chaque année pendant vingt ans. Le compte n'y est pas, alors que les besoins sont énormes. Le plan de relance prévoit certes 2 milliards d'euros supplémentaires sur deux ans pour le parc privé, mais ce montant reste nettement insuffisant pour atteindre les objectifs fixés et faire face à l'élargissement du nombre de bénéficiaires.

une logique purement comptable et complètement aveugle ! Quel est le prix du climat ? Quelle est la valeur des générations futures ? Peut-on parler du retour sur investissement d'un budget qui va dans le sens de la préservation de la vie sur cette planète ?

Au regard des sommes qui ont été engagées pour la baisse des impôts de production- un montant de près de 20 milliards d'euros -, je vous propose, monsieur le ministre, la prise en charge intégrale du coût du chômage partiel. Une telle mesure permettrait de garantir à nos concitoyens qui perçoivent les rémunérations les plus faibles le maintien de leur niveau de pouvoir d'achat et de prévenir l'émergence d'une nouvelle fracture sociale dans notre pays. Pour éviter les effets d'aubaine, seuls les revenus inférieurs à deux fois et demie le SMIC

Je ne développerai pas plus avant sur la nécessité du report modal, si ce n'est pour rappeler qu'à la tonne kilomètre transportée, le rail émet huit fois moins de particules

les locataires modestes du privé étant les plus touchés. Les enjeux écologiques et sociaux liés à la rénovation thermique des bâtiments ont été clairement soulignés par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Les associations déplorent ainsi que le dispositif MaPrimeRénov'reste largement favorable aux ménages les plus aisés au regard d'un reste à charge encore trop

Force est de constater que, malgré les efforts, le compte n'y est pas. C'est pourquoi nous vous proposons d'augmenter fortement les crédits alloués à la rénovation thermique afin d'engager concrètement des moyens à la hauteur de l'ambition affichée- en finir avec la précarité énergétique et les passoires thermiques.

que les obligations fixées par la LOM, en imposant aux collectivités un objectif de 50 % de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène, proportion qui concernerait aussi bien les véhicules particuliers et les utilitaires légers que les véhicules industriels. Il convient de mettre en cohérence les objectifs et les moyens financiers. Tel est

pour la scolarité et l'apprentissage. À la disposition des rectorats, ce fonds permettrait, sur sollicitation des établissements scolaires, de financer

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement souhaite mettre en place une action de rénovation énergétique reposant sur le dispositif MaPrimeRénov'. Les auteurs du présent amendement estiment qu'il serait opportun de renforcer

En prévoyant que les logements seront évolutifs à l'issue de travaux simples, le Gouvernement fait peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte de devoir réaliser des travaux d'adaptabilité.

Compte tenu des enjeux liés au vieillissement de la population, nos politiques publiques doivent permettre à chacun de se maintenir aussi longtemps que possible à son domicile. Il appartient à l'État d'accompagner le financement de l'installation d'équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées afin d'améliorer l'adaptation globale du parc immobilier aux besoins spécifiques de ces personnes.

Guillaume Gontard. Cet amendement vise à créer un fonds de solidarité spécifique aux entreprises corses liées au secteur du tourisme, car l'économie de l'île en dépend. Ce secteur compte entre 8 000 et 11 000 emplois à l'année et pèse 24 % du produit intérieur brut de l'île, hors activité de transport. Les effets délétères du confinement pèsent particulièrement lourd sur l'économie de la Corse, entraînant une baisse d'activité de l'ordre de 35 %. Cette aide qui peut s'ajouter à d'autres mesures de soutien permettrait aux dites entreprises de faire face à leurs charges fixes.

largement rabotées ces dernières années par des politiques injustes et inefficaces. De l'aveu même de la Cour des comptes, ces aides sont un outil puissant de redistribution sociale.

Ce scénario privilégie la mise en oeuvre des priorités de restauration et de modernisation du patrimoine, ainsi que d'amélioration des mobilités du quotidien, pendant une dizaine d'années, à un niveau d'ambition élevé qui s'inscrit en rupture avec les pratiques antérieures.

Il est raisonnable d'anticiper une hausse continue du nombre de collectivités candidates à des financements de l'État. La montée en charge doit donc être à la hauteur. Une enveloppe totale de 500 millions d'euros par an, incluant les 350 millions que nous proposons, permettrait de financer le développement de nouvelles politiques en faveur des vélos, encore trop absentes dans notre pays et pourtant indispensables, à savoir l'accessibilité en gare le réseau cyclable, une offre suffisante de stationnement sécurisé des vélos en gare, l'embarquement des vélos à bord des trains, les services de réparation et de location de vélos dans les gares et une politique éducative les « vélos-écoles » et promue par la fédération des usagers de la bicyclette (FUB). L'enjeu est culturel et éducatif. Il s'agit de réduire les tensions qui résultent de l'irruption forte des vélos sur un territoire jusqu'ici presque exclusivement dévolu aux véhicules motorisés et déjà compliqué pour les piétons.

21 % de nos concitoyens disaient rencontrer des difficultés pour se procurer une alimentation saine, leur permettant d'assurer deux repas par jour. Cette situation n'a fait qu'empirer. Les associations caritatives tirent le signal

en février dernier, le besoin de financement global pour gommer le retard d'investissement et éviter des fermetures de lignes est évalué par SNCF Réseau

des protocoles avec les régions, alors qu'il ne sera pas en mesure de les respecter, faute de crédits pour éviter la fermeture de ces 9 000 kilomètres

1,5 milliard d'euros, soit 150 millions annuels, l'investissement nécessaire d'ici à 2030 pour créer quinze nouvelles lignes nationales.

Il est cependant possible d'atteindre ces objectifs sans surcoût final, comme l'ont montré de nombreux exemples locaux, pour lesquels le prix à l'assiette est identique. La transition nécessite temporairement des moyens pour structurer des circuits d'approvisionnement locaux, sensibiliser les personnels, réaliser des diagnostics, en particulier sur le gaspillage alimentaire, ou encore financer des investissements matériels. matériels. Cet amendement vise à financer ce surcoût temporaire qui permet l'enclenchement d'une boucle vertueuse, puisque, la réduction du gaspillage et le travail de produits bruts, locaux et de saison, les restaurants réalisent des économies qu'ils peuvent réinjecter dans l'achat de produits bio et de qualité. Si cette proposition, qui consiste à accorder des moyens aux collectivités pour la mise en oeuvre de la loi Égalim, a été en partie reprise dans le plan de relance, le soutien apporté par l'État dans le budget actuel est loin d'être suffisant. Cet amendement a donc pour objet d'augmenter les financements prévus

je vous remercie,

Comme lors du PLFR 4, nous proposons de mettre en place un fonds d'aide à la quittance pour épauler les locataires les plus fragilisés par la crise qui ne parviennent plus à payer leur loyer. L'augmentation prévisible du chômage nécessite des mesures fortes pour empêcher les Français de basculer dans la précarité. L'urgence est d'aider les personnes fragilisées par la crise à conserver leur logement. On sait en effet que le logement représente les deux tiers de la consommation préengagée des ménages pauvres. Le plan de relance ne signifie pas la sortie de la crise. Il doit s'accompagner de mesures d'urgence renforcées pour éviter qu'une crise sociale durable ne s'installe. Cette urgence sociale est relayée depuis des mois, non seulement par les acteurs de la solidarité, mais aussi par les bailleurs sociaux et les associations d'élus.

ce fonds n'est pas universel. Il est destiné aux personnes en situation de précarité sociale et reste ouvert selon les critères préalablement définis par chaque département. Les bailleurs sociaux veillent à soutenir leurs locataires en difficulté de paiement. Le mouvement HLM et les associations nationales de locataires ont signé une charte en faveur des locataires en situation de fragilité économique pendant la crise du covid-19. Les informations manquent quant à la situation dans le secteur privé. Cet amendement a pour objet d'abonder le FSL pour gérer l'aide d'urgence à la quittance. La gestion de cette aide pourra être assurée par une cellule d'urgence « crise sanitaire » créée au sein du FSL. Cette cellule viendra en aide aux locataires du parc locatif social ou privé, ayant subi une perte de revenus à cause de l'épidémie et se trouvant en difficulté

à M. Jacques Fernique. Cet amendement propose un renforcement exceptionnel de la prime à la conversion automobile, mais en faveur des mobilités douces. Ainsi, il est proposé d'élargir le champ d'utilisation de la prime à la conversion et de réserver 150 millions d'euros à une prime destinée aux personnes ne rachetant pas de voiture, une prime pour abandon de véhicule. Pour atteindre les objectifs climatiques et lutter efficacement contre la pollution de l'air, il est indispensable de réduire l'usage de la voiture individuelle, en proposant à nos concitoyens un panel de solutions alternatives plus propres. Cette prime permettra de financer l'acquisition d'un vélo, vélo électrique ou vélo-cargo, un abonnement aux transports en commun ou encore un abonnement à un service d'autopartage ou de covoiturage.

plus respectueux de l'environnement et moins consommateurs de ressources. Du fait de la crise économique, l'investissement des entreprises industrielles risque d'être sacrifié. Leur encours de crédit a augmenté de 13 % sur l'année. Elles ont réduit dans le même temps leurs dépenses d'investissement d'environ 14 %. Pourtant, l'enjeu de modernisation de l'industrie française est plus pressant que jamais face au double défi de la compétitivité et de la transition environnementale. La mission « Plan de relance » prévoit plusieurs dispositifs d'aides à l'investissement, notamment dans la robotisation ou la rénovation énergétique des bâtiments. Cependant, le soutien au « verdissement » des procédés et des produits industriels eux-mêmes apparaît sous-dimensionné. Sur les 500 millions d'euros prévus en autorisations d'engagement pour l'économie circulaire, seuls 84 millions pourraient être dépensés en 2021 dans le cadre d'actions de long terme menées par l'Ademe.

Économie circulaire et circuits courts, du programme 362, « Écologie ». Il s'agit de mettre en place un dispositif plus souple et plus rapidement mobilisable de guichet de cofinancement des investissements industriels, afin de développer l'écoconception des produits, l'économie de ressources dans les procédés, la réduction de l'usage du plastique et la réduction des déchets. Quel

j'imagine que l'intention du rapporteur spécial était d'abord de faire avancer sa proposition, et non de retirer des crédits à cette

baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, soit- je crois -l'équivalent d'un peu plus de 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires ... Pour parler comme Julien Bargeton, j'eusse aimé que vous vous laissassiez tenter ... aurions ainsi dégagé des marges supplémentaires pour financer un plan de relance et un plan d'urgence qui, s'ils ont le mérite d'exister, ne couvrent pas l'intégralité du champ des besoins, comme le montrent tous ces amendements.

les lois de programmation des finances publiques, les recommandations de la Cour des comptes, les avis du Haut Conseil des finances publiques, les marchés financiers, l'article 40 de la Constitution, les contraintes européennes- on l'a vu cette semaine avec la TVA -, les sanctions éventuelles de l'Union européenne- 0,2 % du PIB -, les commissions mixtes